la position du Gouvernement, qui comporte trois points. Premièrement, le texte du Gouvernement, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, insérait dans le code pénal une disposition interprétative sur les notions de contrainte et de surprise

raisons. D'abord, étant interprétatif, il s'appliquera immédiatement. Tous les mineurs, y compris ceux qui auront été victimes de violences sexuelles dans le passé, pourront en profiter. Ce texte ne crée donc pas un double régime qui s'appliquerait dans les décennies à venir.

En indiquant que la contrainte est caractérisée en cas d'abus de la vulnérabilité d'un mineur de quinze ans ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel, la loi aura nécessairement pour conséquence pratique, pour les mineurs les plus jeunes,

La loi ne peut pas fixer ces âges, mais nous pourrons le rappeler dans une circulaire, en faisant état notamment des débats tenus devant le Parlement.

mais, comme l'a indiqué le Conseil d'État, des difficultés se posent de nature constitutionnelle et conventionnelle. En effet, instituer une présomption de culpabilité, même simple,

caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». D'une part, dès lors qu'il y a abus de la vulnérabilité et absence de discernement, la contrainte ou la surprise sont nécessairement caractérisées. Prévoir, comme l'a fait la commission des lois, qu'elles « peuvent être » caractérisées serait, me semble-t-il, source d'ambiguïtés. D'autre part, il me semble important de préciser qu'il s'agit du discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel, et non du discernement dans l'absolu. Cette formulation protège mieux le mineur, qui peut avoir un discernement suffisant dans d'autres domaines.

les délégations aux droits des femmes des deux assemblées, en concertation avec les associations de victimes, de lutte contre les violences sexuelles et de protection de l'enfance, soulignent avec force que l'expression « maturité sexuelle suffisante » est à proscrire.

d'une mineure de moins de quinze ans puisse être suffisante, cette rédaction affaiblit significativement la portée de l'appréciation de la notion de contrainte, que ses promoteurs se proposent pourtant d'amplifier. Elle implique qu'une maturité sexuelle suffisante d'une enfant ou d'une adolescente de moins de quinze ans pourra être invoquée par la défense afin de nier la responsabilité d'un adulte dans le cadre d'un viol ou d'une agression sexuelle. Cette terminologie renforce donc la probabilité pour les auteurs présumés d'infractions à caractère sexuel sur mineur de quinze ans d'être acquittés ou de voir leur peine réduite bien en deçà de l'infraction commise. commise. Pour être on ne peut plus clairs, nous considérons que les arguments tels que : « elle a l'air d'avoir seize ans », « elle a essayé de me séduire par son comportement », « elle porte des tenues courtes », « elle prend des dans des positions suggestives », etc., s'ils sont bien bel et bien légitimes du point de vue du défendeur et de la garantie des principes des droits de la défense, doivent être combattus sur le terrain politique et faire l'objet d'une condamnation sociale forte. Cette condamnation sociale, qui s'est fortement exprimée lors des affaires de Pontoise et de Melun, doit être encouragée et non pas piétinée par le fait d'insérer dans le code pénal l'existence d'une maturité sexuelle suffisante des mineurs de quinze

Je sais bien que cette matière est vraiment difficile et, en réalité, on se rend compte qu'elle est compliquée. Il ne s'agit pas ici de la principale innovation

lui permettre d'avoir des références : il reste libre de décider qu'il y a eu contrainte morale ou pas. pas. Nous ne voulons pas revenir au texte du Gouvernement. Madame la garde des sceaux, je vous ai vraiment écoutée avec beaucoup d'attention et je reconnais toute la valeur du point de vue

capacité d'examiner individuellement chaque affaire en fonction de la réalité de la situation qui lui est soumise. Je vous en conjure, faisons quand même confiance au juge, dès lors que la loi est suffisamment précise. Permettez-moi

prudente, ne constitue pas un pas en avant fort avec une modification de la charge de la preuve, afin que le coupable puisse être plus facilement condamné et que la victime ne voit pas peser sur elle une contribution à la démonstration de la culpabilité de son agresseur, ce qui la conduirait à devoir se justifier. Or ce n'est vraiment pas un état d'esprit convenable pour punir les agresseurs de mineurs.

revient à affirmer dans le texte de la commission que la simple minorité de quinze ans caractérisera la contrainte, donc le viol ou l'agression sexuelle, sans appréciation par le juge. Cela me semble évidemment excessif. C'est, me semble-t-il, uniquement si le mineur de quinze ans n'a pas le discernement suffisant que l'on pourrait parler de viol.

ce que les auxiliaires de justice ou les magistrats- je n'ose parler des auteurs ou des victimes -comprendront du régime juridique applicable

redoutables, veut imposer le critère de « maturité sexuelle suffisante », ce que je trouve, je le dis, terrifiant. Pas moi ! Je n'ose imaginer les débats devant les juridictions pénales au cours desquels il faudra évaluer, quelques années après les faits, la maturité sexuelle de la victime. Eh oui ! Si tout le monde ici souhaite que l'on simplifie le sort des victimes et que l'on fasse en sorte

madame la secrétaire d'État, le Président de la République, le 25 novembre dernier, au cours d'un discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, indiquait, justement à propos des affaires que l'on a citées : « Je veux ici vous donner une conviction personnelle : nous devrions sans doute aligner sur l'âge de la majorité sexuelle, fixée dans le droit à quinze

vous n'y arrivez pas, et vous oubliez complètement que, devant la cour d'assises, c'est l'intime conviction qui est importante, et non pas la motivation juridique. Les questions qui ont été évoquées devant les assises et qui ont notamment abouti à des acquittements concernent précisément la notion d'intime conviction. Je comprends maintenant pourquoi vous envisagez dans le projet de loi sur la justice la création d'une juridiction

vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » On parle là de faits qui sont commis sur la personne d'un mineur ou d'une mineure de quinze ans. Cela signifie que l'on considère que des mineurs

ou de dix-neuf ans. On se trouve là dans un cas de figure où la différence d'âge n'est pas significative et où il n'y a pas d'autorité de droit ou de fait exercée sur la victime. Notre troisième critère alternatif vise vraiment à couvrir le maximum de situations, voire toutes les situations.

Le scrutin est ouvert.

inspirés par les enquêtes de terrain réalisées par les membres de cette instance et de cette association, vise à préciser à la fois le caractère éventuellement psychologique des violences, l'étendue des formes de pression pouvant être constitutives de menaces, en y incluant le caractère coercitif d'un environnement- on pense au bizutage au cours duquel des jeunes filles ou des jeunes garçons peuvent se retrouver dans des situations où ni le consentement ni le non-consentement n'ont pu être identifiés et qui sont déterminés par l'environnement -, et la prise de conscience des stratégies tendant à tromper la victime. Il s'agit ici de préciser le respect du consentement. J'y insiste, cet amendement est

? Cet amendement vise à inscrire dans la loi des clarifications concernant les éléments constitutifs des agressions sexuelles, notamment du viol, mais il est mal rédigé. En effet, ce type de dispositions visant à interpréter des notions de droit pénal La jurisprudence n'a d'ailleurs pas besoin de ces précisions : l'analyse de la jurisprudence récente démontre bien la prise en compte des violences psychologiques par les juridictions. De il nous semble maladroit de renvoyer aux violences psychologiques délictuelles prévues par d'autres articles du code pénal, la notion de violence psychologique pour l'exercice d'un viol étant plus large et détachée d'une attraction particulière. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère Madame la garde des sceaux,

parole est à Mme Michelle Meunier. Actuellement, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Or les termes « commis sur » posent problème. En effet, si un adulte force un enfant à lui faire une fellation, le droit considère qu'il s'agit d'un viol, car il y a eu pénétration du sexe de l'adulte dans la bouche de l'enfant. Si cet adulte fait une fellation de force à un enfant, les juges considèrent qu'il s'agit d'une agression sexuelle, car l'introduction du sexe de l'enfant dans la bouche de l'adulte n'est pas reconnue comme une pénétration commise sur le mineur. Malgré les séquelles psychologiques identiques

En effet, la définition du viol a déjà été modifiée par la commission des lois, afin de réprimer comme des viols, et non comme des agressions sexuelles, les actes de pénétration sexuelle forcés, mais sur la personne de l'auteur. La commission a précisé que le viol pouvait être caractérisé par des actes de pénétration sexuels commis, tant sur la personne d'autrui que sur la personne de l'auteur. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu'il ait été réalisé sur la victime ou non, sera considéré comme un viol. Ainsi, les faits de fellation forcés que vous décrivez sont déjà couverts par l'alinéa 7 de l'article 2 du texte de la commission. Néanmoins, la

d'instaurer une présomption, même simple, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui protègent la présomption d'innocence. Les seules présomptions admises par notre droit, de manière exceptionnelle, concernent la matière contraventionnelle ou délictuelle et prévoient, à chaque fois de façon très précise, les conditions permettant de les écarter. Par ailleurs, la présomption qui est proposée par votre commission s'appliquerait, soit pour des mineurs incapables de discernement, ce qui constitue une hypothèse juridique claire, même si elle est difficile à prouver dans certains cas, soit

En pratique, que signifiera l'existence d'une présomption devant la cour d'assises ? Faudra-t-il que la cour et les jurés répondent à une question supplémentaire sur l'existence éventuelle d'une différence d'âge significative entre l'auteur et la victime ?

Quelles seront enfin les conséquences de la présomption sur l'exigence de motivation ? Bref, vous m'aurez comprise, il me semble que l'on ne peut pas construire une présomption, avec les conséquences graves que cela entraîne, à partir d'une définition juridique aussi floue que celle

sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à celui qui introduit dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Le présent amendement tend à compléter l'article l'article 222-23 du code pénal, qui définit le viol. Il précise ainsi que la contrainte, qui constitue l'un des critères du viol, est nécessairement constituée quand l'auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de treize ans. Il marque ainsi l'interdiction d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant. Ce seuil de treize ans a été retenu par cohérence avec le droit pénal, qui fixe la responsabilité pénale des mineurs à cet âge. Il permet par ailleurs de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescents et des adolescentes d'une quinzaine d'années et de jeunes majeurs et d'éviter que ces derniers ne se retrouvent accusés de viol. J'ajoute qu'au Royaume-Uni, pays qui n'est pas réputé bafouer les droits de la défense, un enfant de moins de treize ans n'a

un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte. Les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l'article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes. Cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime, qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l'agression sur la victime. Or il revient aux adultes de protéger les enfants, et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il est inacceptable que, en raison de cette subjectivité inhérente à la définition pénale du viol, les mêmes faits, dans des circonstances similaires, puissent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l'ont montré de récentes affaires. Il est essentiel que la loi affirme « l'interdiction absolue d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l'interdit constituant un crime ». Je rappelle que la solution consistant à créer un seuil d'âge pour marquer un interdit n'est pas sans précédent : l'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, qui constitue un délit, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure, et non comme une présomption d'absence de consentement. L'atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, de contrainte, de violence ou de surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime. La même logique pourrait s'appliquer pour les relations sexuelles avec un mineur de moins de treize ans et un adulte. L'élément intentionnel de l'infraction résulterait de la pénétration sexuelle elle-même. Posons-nous la question : peut-il y avoir des pénétrations sexuelles involontaires, comme il y a des homicides involontaires ? Il ne peut y avoir de pénétration sexuelle par hasard. Il résulterait aussi de la connaissance de l'âge de la victime par l'auteur des faits. Pour se défendre, celui-ci aurait la possibilité de prouver qu'il ne connaissait pas l'âge de la personne. Les droits de la défense seraient donc respectés. Je rappelle que, il y a peu, cette assemblée était largement hostile à l'allongement des délais de prescription. Aujourd'hui, ces dispositions font majoritairement consensus. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour la fixation d'un seuil en deçà duquel un rapport sexuel entre une personne majeure et un enfant sera considéré comme un crime. D'ici là, combien d'entre eux devront en payer le prix ? La parole

comme le faisait très justement remarquer le rapport de nos collègues députés Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain, au nom de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, marque la limite indiscutable de l'enfance. Qui oserait décemment affirmer

Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d'avoir un rapport sexuel avec un adulte. » Jusqu'à quel âge est-on encore un enfant ?

de treize ans. Le procureur Molins, désormais promis à de nouvelles fonctions très importantes, a lui-même indiqué, lors de son audition à l'Assemblée nationale, qu'il lui paraissait cohérent d'instaurer ce seuil.

n° 130 du Gouvernement. L'introduction d'une présomption de culpabilité, même simple, en matière criminelle porte atteinte au principe constitutionnel de présomption d'innocence, mais cette atteinte est proportionnée à l'objectif d'intérêt général que l'on cherche à atteindre, à savoir la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. La définition de notre présomption de contrainte nous semble donc répondre aux exigences constitutionnelles.

et 105, qui visent à créer une présomption de contrainte en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans. Cette disposition pose plusieurs difficultés. En fragmentant le régime de protection des mineurs, l'adoption de ces amendements aurait pour conséquence de moins protéger les mineurs de treize à quinze ans. Ce risque a d'ailleurs été souligné par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants. Ce risque a également été souligné par des représentants de la chambre criminelle. L'introduction d'un « âge seuil » risque également d'être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple, pour l'application de la notion de contrainte morale. La création d'une telle présomption ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l'existence d'une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ou L'instauration d'une présomption de non-consentement en deçà de treize ans instaurerait une zone grise quant à la répression pénale de ces comportements, qui pourraient inciter à se reposer

Aujourd'hui, en raison de la majorité sexuelle fixée à quinze ans, les mineurs de quinze ans bénéficient d'une protection particulière. Les circonstances aggravantes dépendent également de la minorité de quinze ans. Introduire un deuxième seuil d'âge reviendrait à affaiblir ce seuil de quinze

Le Sénat s'est déjà prononcé sur cette question lors du vote de la proposition de loi de notre collègue Philippe Bas en mars dernier. La création d'un seuil d'âge de criminalisation paraît simple et évidente. Néanmoins, il est inopérant et contre-productif de fragmenter les régimes de protection des mineurs en fonction d'un seuil d'âge. Il est préférable de privilégier une appréciation concrète de chaque situation plutôt qu'une automaticité. La proposition de loi adoptée par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineures, quel que soit leur âge. L'introduction d'un seuil d'âge ne protégerait qu'une partie d'entre elles. Pourquoi retenir une telle solution inégalitaire ?

d'une date d'anniversaire, et donc d'un seuil d'âge. Comme l'a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l'âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu'il est aujourd'hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien. Bien sûr ! Surtout, une telle disposition est manifestement contraire à la Constitution. Je fais miens les arguments de Mme le garde des sceaux et du président Philippe Bas sur l'inconstitutionnalité d'une telle disposition. Aujourd'hui, au regard des enquêtes de sexualité réalisées en France, il est parfaitement envisageable d'imaginer une adolescente de douze ans et demi,

au-delà de la majorité du partenaire le plus âgé qualifierait automatiquement de crime, et non pas de délit comme actuellement, un tel comportement. On ne peut pas prendre le risque d'une telle injustice. Ce n'est vraiment pas possible ! Quel est l'avis du Gouvernement

et conventionnelles que j'ai eu l'occasion d'exposer devant vous. J'ajouterai simplement que, en matière criminelle, le principe de la présomption d'innocence paraît interdire l'instauration d'une présomption, même simple,

pour l'âge de treize ans, cela précarise la situation des mineurs de plus de treize ans, pour lesquels, en quelque sorte, sera posée implicitement par le législateur une présomption de consentement, ce qui sera évidemment invoqué par la défense. Si, comme il résulte du texte, la présomption n'est pas présentée comme irréfragable, un débat sera en tout état de cause toujours possible sur l'existence ou non de la contrainte. En outre, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer en défendant l'amendement de suppression, on ne sait pas comment, d'un point de vue procédural, l'existence d'une présomption sera prise en compte devant une cour d'assises, tant au regard de la procédure et des questions à la cour qu'en ce qui concerne l'exigence de motivation. une telle disposition, par nature plus sévère, ne pourrait s'appliquer, je l'ai déjà dit, immédiatement aux faits commis avant la nouvelle loi, à la différence de la disposition interprétative que nous proposons.

des règles spécifiques pour les mineurs de treize ans, car la fixation d'un double seuil d'âge- quinze ans pour préciser les notions de contrainte et de surprise ; treize ans dans d'autres cas -aboutirait à une réforme particulièrement complexe, assez peu lisible et compréhensible pour l'opinion publique. Surtout, la fixation d'un seuil de treize ans donnerait, à tort, bien sûr, l'impression qu'une atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur plus âgé serait plus plus ou moins licite, ce qui n'est évidemment pas acceptable. À mon sens, un seul et unique seuil doit être fixé par le code pénal : c'est celui qui existe déjà, c'est-à-dire quinze ans.

par ma collègue Laurence Cohen, visent à instaurer un seuil d'âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte serait un crime, passible de vingt ans de réclusion criminelle. Il s'agit de créer un crime autonome de celui de viol et de sortir ainsi de la question du consentement et des définitions, parfois sujettes à caution, des critères de « violence, contrainte, menace ou surprise Cette proposition correspond à la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes ; elle est également portée par de nombreuses associations de lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants. de mon appréhension quand il s'agit de créer de nouvelles infractions et de mon aversion naturelle pour le mouvement qui conduit à l'instauration d'une justice d'exception

par les affaires de Meaux et de Pontoise, les affirmations, souvent fausses, qui ont été relayées auprès de nos concitoyens et les débats, parfois très violents, qui ont eu lieu depuis quelques mois m'ont convaincue d'une chose : il faut faire preuve de pédagogie auprès de nos concitoyens afin qu'un débat serein puisse avoir lieu. Si, selon un récent sondage IPSOS, 81 % des Français sont favorables à ce que la loi prévoie un seuil d'âge minimum en dessous duquel un acte de pénétration sexuelle commis par une personne majeure serait automatiquement considéré comme un viol, on ne peut balayer cela d'un revers de main.

Marie-Pierre Monier, pour explication de vote. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que nos débats doivent permettre d'aboutir à un texte qui devra, avant tout, protéger les mineurs victimes de viol en fixant un interdit suffisamment fort, qui serve à la fois à la pénalisation des auteurs et à la prévention.

plutôt que comme victimes d'un délit. L'article 121-3 du code pénal dispose, dans son premier alinéa, qu'« il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », en conséquence de quoi la caractérisation de l'infraction à la loi en matière d'agissements sexuels reconnaît reconnaît le caractère intentionnel. Ce point n'est donc pas l'objet de débat ; il reste à préciser les termes juridiques qui permettront une application harmonieuse du code pénal sur l'ensemble du territoire. Le texte qui sera issu de nos débats doit laisser le moins de prise possible à la subjectivité. Pour cela, il doit définir l'acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de treize ans comme un crime. C'est à cette condition seulement que l'acte sera passible des mêmes sanctions que celles prévues en cas de viol, sans que les critères de violence, contrainte, menace ou surprise définis par l'article 222-23 du code pénal soient pris en considération et sans que puisse être évoquée la question du consentement de la victime. la question du consentement de la victime. Aucune règle au niveau européen ne s'oppose à l'adoption d'une telle proposition, puisqu'une telle mesure existe déjà au Royaume-Uni ou encore en Belgique. L'adoption de l'amendement n° 24 rectifié de l'amendement n° 24 rectifié créera une nouvelle incrimination pénale spécifique, celle de crime de violence sexuelle sur enfant, posant l'interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un enfant, comme le recommande notamment le Conseil national de la protection de l'enfance. C'est le moyen le plus efficient pour poser un interdit clair à destination des adultes. La parole est à M.

où il est écrit que beaucoup de pathologies sont les conséquences de violences sexuelles vécues dans l'enfance : le diabète, l'hypertension, certains cancers, l'endométriose

la violence sexuelle détruit l'humanité, car elle est la racine de la plupart des faits de violence extrême, y compris d'actes de terrorisme. Il faut la combattre clairement et protéger les enfants, qui en sont les premières victimes.

demande de juger une affaire qui aurait pu être qualifiée de viol pour ne pas aller devant la cour d'assises, car il a la certitude que, devant le juge professionnel, il obtiendra une condamnation qu'il risque de ne pas obtenir devant la cour d'assises. Qui sont les juges de la cour d'assises ? Ce sont ceux qui nous élisent Ont-ils moins de clairvoyance lorsqu'ils élisent leurs représentants que lorsqu'ils jugent ? Que craignez-vous de ces juges ? Ce sont eux qui ont la totale légitimité.

nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui est le point fondamental. Heureusement, Mme la rapporteur a fait inscrire au tout début de notre texte un certain nombre

vous avez défendu les alinéas 8 et 9, qui disposent que la contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis. Vous défendez donc un projet dans lequel la contrainte est présumée et vous nous dites après, contre nos amendements, qu'il ne peut pas y avoir de présomption. Ce n'est pas cohérent ! Nous devons

Celle du Gouvernement, qui simplifiait la preuve du viol, en disant que l'abus de la vulnérabilité pouvait être une preuve de la surprise,

dont il peut s'adjoindre les services, le soin de déterminer si la jeune fille ou le jeune garçon qui a été victime d'agression savait exactement ce qu'il faisait ou en avait conscience. Le magistrat

en quelques mois. Il a rendu public un rapport d'information de plus de 130 pages, après avoir procédé à l'audition de 64 personnalités- monde associatif, médecins, juristes, représentants des administrations, magistrats, avocats -et à dix déplacements, pour se rendre compte sur place des problématiques.

existe déjà un seuil à quinze ans. Pourquoi, monsieur Sueur ? Je vais vous redire ce que nous ont expliqué les magistrats- nous en avons auditionné de très nombreux -et le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; je pense qu'il sait de quoi il parle. L'introduction d'un seuil d'âge d'être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple pour l'application de la notion de contrainte morale. Une telle disposition ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l'existence d'une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de quinze L'instauration d'un seuil d'âge instaurerait cette fameuse zone grise quant à la répression pénale de ces comportements, qui pourraient inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d'atteinte sexuelle et donc à mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

Avis défavorable. La création d'une circonstance aggravante au délit d'atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l'âge de treize ans. L'âge clé dans la protection des mineurs doit rester l'âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d'autre seuil d'âge, au risque d'affaiblir le régime actuel de protection des mineurs. C'est de l'entêtement

sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, pour mieux accompagner les victimes, qui peuvent se retrouver démunies devant la complexité des procédures, des associations d'aide aux victimes devraient pouvoir les accompagner à tous les stades de la procédure. Aujourd'hui, le mineur peut être accompagné de son représentant légal, mais celui-ci peut être concerné par les faits. De plus, le code de procédure pénale prévoit qu'il n'est possible de désigner un administrateur que que lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. Le mineur doit donc recevoir l'aide d'une association entre le dépôt de plainte et l'aboutissement de la procédure. Quel

M. Gérard Poadja. Cet amendement vise à systématiser l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'atteinte sexuelle et d'agression sexuelle. Ce fichier de sûreté contient les identités et les adresses des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs ou de crimes violents. Il permet aux forces de l'ordre de localiser rapidement ces individus et facilite les enquêtes. À ce jour, l'auteur d'une atteinte sexuelle ou d'une agression sexuelle n'est pas automatiquement inscrit dans ce fichier, contrairement aux auteurs de viol puisque les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans échappent à l'automaticité de l'inscription. L'inscription ou non dans ce fichier relève de la décision d'un juge. Je tiens à rappeler ici que je ne remets nullement en cause la capacité d'un juge à décider d'une telle mesure. Cependant, il n'est pas acceptable que des personnes condamnées pour de telles infractions ne soient pas référencées afin de pouvoir prévenir de tristes récidives. Chaque année, près de 62 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol en France, ce qui représente 44 % des crimes commis. Le taux de récidive en 2017 était de 5 % pour les crimes de viol et de 23 % pour les délits sexuels. Quel l'avis de la commission ? Cet amendement vise à prévoir l'inscription automatique des délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle au motif que, contrairement aux viols, ces délits ne feraient pas l'objet d'une inscription automatique. Cette interprétation est fausse : l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-2 prévoit bien que seuls les délits punis d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement ne font pas l'objet d'une inscription, sauf décision contraire de la juridiction.

Cohen ! Le juge criminel, comme ce doit toujours être le cas en matière pénale, conservera un pouvoir d'individualisation de la peine. Très grande clarification, très grande fermeté,

Le scrutin est ouvert.